l'amendement n° 19. Nous demandons la suppression de l'article 9, qui prévoit le transfert aux régions volontaires du matériel roulant appartenant à SNCF Mobilités. En effet, ce matériel est le plus souvent en mauvais état et un tel transfert constituera une charge supplémentaire pour les régions, qui devront notamment assurer seules son renouvellement. ce transfert participe du dépeçage de l'entreprise historique et organise son affaiblissement. Cette possibilité, déjà offerte par la loi portant réforme ferroviaire, semble donc contestable. En effet, les régions sont exsangues du fait de la baisse des dotations et elles ont déjà fait des efforts très importants pour développer l'offre ferroviaire. Les transports sont devenus le premier poste de dépense des régions. Cet effort supplémentaire qui leur est demandé ne paraît donc pas acceptable, ouverture à la concurrence ou non,

En effet, les régions n'ont pas à supporter les conséquences financières de décisions prises antérieurement à la régionalisation du transport ferroviaire. Le législateur doit également résoudre la question de la refacturation de la TVA ayant été déduite par SNCF Mobilités lors de l'achat du matériel appartenant dorénavant aux régions.

pour présenter l'amendement n° 53. Le matériel roulant, les ateliers de maintenance, les gares, au même titre que les services considérés comme d'intérêt commun, font partie de ce que les économistes appellent les « facilités essentielles

des transports, l'AOT, qui les mettait à la disposition de SNCF Mobilités. Cet article vise à réaffirmer le caractère automatique du transfert de matériels lorsque l'AOT en fait la demande.

on a de bonnes raisons de penser qu'elles choisiront les matériels les plus performants. Si SNCF Mobilités perd des contrats au profit de nouveaux concurrents, que deviendront les trains en surplus ? Certains seront sans doute encore tout à fait performants et susceptibles de rouler ; qui les entretiendra

Je rappelle que cette disposition ne fait que renforcer une mesure qui avait été introduite dans la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, et qu'il s'agit d'une simple possibilité offerte aux régions, et non d'une obligation. Les régions ont investi plus de 11 milliards d'euros, entre 2011 et 2015, pour renouveler plus de 80 % du matériel roulant ; il me semble donc normal qu'elles puissent en récupérer la propriété si elles le souhaitent. Je ne serais pas opposé à ce qu'on précise le dispositif, si cela s'avérait nécessaire, pour évoquer les questions précises posées par les auteurs de ces amendements, mais la suppression de l'article équivaudrait à un recul, puisqu'une disposition de cet ordre existe déjà dans le code des transports. Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis sera défavorable.

De plus, les régions n'ont pas demandé à devenir propriétaires de ces ateliers de maintenance, dont le coût de rachat est non négligeable. Nous demandons donc la suppression de cet article, qui instaure une charge nouvelle non compensée pour les régions et qui affaiblit l'entreprise historique, pour créer des conditions favorables à l'arrivée sur le marché de nouveaux opérateurs.

Cet article prévoit le transfert automatique des ateliers de maintenance utilisés par SNCF Mobilités aux AOT lorsque celles-ci en font la demande. Sur le principe, nous ne sommes pas défavorables à cette disposition, réclamée par les régions. Si les ateliers de maintenance sont aussi considérés comme étant des facilités essentielles, leur accès doit être libre pour toutes les entreprises ferroviaires ; le transfert de leur propriété aux AOT devrait permettre d'assurer ce libre accès.

Dès lors, comment penser ce transfert ? Souhaitez-vous créer des ateliers partagés ? À la lumière de ce constat, ne serait-il pas possible d'envisager d'autres hypothèses, comme le transfert de ces établissements de maintenance et commercial SNCF Réseau ? Certaines organisations le proposent, en tout cas, et, dans la perspective d'une réflexion globale sur les mobilités, cette hypothèse n'est pas dénuée d'intérêt. Nous avons aussi quelques interrogations sur l'avenir de certains centres de maintenance.

Par ailleurs, certains ateliers de maintenance ont anticipé le tassement de leur activité, lié au fait que le matériel roulant est assez neuf et demande aujourd'hui peut-être moins d'entretien qu'hier. Certaines nouvelles technologies permettent par exemple un entretien plus facile et plus rapide grâce au recours

et si le contrat d'exploitation des TER est remporté par un concurrent de SNCF Mobilités, il semble plus logique que ce soit la région qui en soit propriétaire et en assure l'accès au nouvel opérateur, plutôt que SNCF Mobilités. figure d'ailleurs parmi les recommandations présentées par l'ARAFER dans sa contribution intitulée « Lever les obstacles pour une ouverture à la concurrence réussie ». En ce qui concerne les inquiétudes relatives aux charges entraînées par ce transfert pour les régions,

En revanche, transférer Gares & Connexions à SNCF Réseau, avec tous les moyens adéquats, sous la forme d'un service doté d'autonomie comptable, s'inscrirait dans la continuité naturelle qui existe entre les activités de gestion du réseau et de gestion des gares.

De même, l'accès aux gares est, pour les différents utilisateurs du système ferroviaire, une interface nécessaire entre la ville et l'accès à la mobilité ferroviaire dans sa dimension de service ouvert au public. Il existe donc une continuité naturelle entre les activités de gestion du réseau et de gestion des gares. Techniquement, la gestion de l'affectation des voies aux trains, la gestion des quais et le pilotage de l'information des voyageurs

cette disposition purement idéologique aura pour conséquence la sortie des gares et des infrastructures du domaine public. L'Union européenne ne nous oblige ni ne nous invite à emprunter cette voie ultralibérale. Les gares sont des outils d'aménagement du territoire et n'ont pas vocation à être exploitées selon une logique comptable pour réaliser des bénéfices. Il nous semble évident que le projet de filialisation de Gares & Connexions a pour finalité de permettre à terme la vente de gares, ce qui aura immanquablement pour effet d'entraîner la disparition progressive de nombreuses dessertes jugées non rentables et un affaiblissement dramatique du maillage du territoire. Pour des raisons tant sociales qu'écologiques, l'adoption d'une telle disposition serait catastrophique.

notamment le fait que sa mise en oeuvre « nécessiterait un contrôle accru du régulateur sur les flux entre Gares & Connexions et le reste de l'EPIC concerné » et qu'elle « ne lèverait pas totalement la suspicion quant à l'indépendance de Gares & Connexions, le président de l'EPIC

Pourtant, séparer le gestionnaire de gares de SNCF Mobilités, opérateur historique de transport, est impératif pour assurer le respect des règles concurrentielles et garantir l'accès de toutes les entreprises ferroviaires aux gares dans des conditions d'équité. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État a d'ailleurs indiqué que la solution retenue dans celle-ci permettrait une mise en conformité avec le droit européen. Pour répondre aux inquiétudes légitimes des auteurs de ces amendements, je rappellerai que l'article 11 prévoit que l'État soit détenteur de 100 % du capital social de Gares & Connexions au moment de sa transformation en société anonyme et qu'il demeure en tout état de cause actionnaire majoritaire. Il n'y a donc pas de privatisation des gares. L'ouverture du capital social à d'autres investisseurs permettra d'investir dans le développement

du Gouvernement ? Nous sommes tous d'accord sur le fait que le rattachement actuel de Gares & Connexions à SNCF Mobilités pose problème dans la perspective de l'ouverture à la concurrence. réfléchir à son positionnement dans ce nouveau contexte. Je veux insister sur l'importance des gares au regard de la fiabilité et de la régularité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 de problèmes de fiabilité des installations. Il s'agit d'un enjeu majeur en termes de transport ferroviaire. J'en suis convaincue, il faut absolument simplifier la répartition des actifs

gares. Je pense à l'inscription des gares dans la ville, bien sûr, au développement des services que les voyageurs peuvent souhaiter trouver sur leur trajet. Je souhaite également insister sur l'importance de l'intermodalité et le rôle que les gares doivent jouer dans une politique

Les économistes qui théorisent l'utopie d'un marché authentiquement libre et d'une concurrence non faussée proposent en effet que les facilités essentielles soient gérées d'une manière totalement neutre.

les auteurs de cette proposition de loi indiquent qu'il s'agit de « garantir un accès transparent et non discriminatoire des entreprises ferroviaires aux gares de voyageurs ». Une telle démarche permettrait d'offrir « une indépendance organisationnelle et fonctionnelle vis-à-vis

? Cet amendement vise à rattacher Gares & Connexions à SNCF Réseau, en tant que direction dédiée, plutôt que d'en faire une filiale de l'EPIC de tête.

Comme vient de le rappeler M. le président de la commission, le rattachement de Gares & Connexions à SNCF Réseau semble à première vue aller de soi, puisqu'il permettrait de réunifier la gestion du patrimoine des gares, qui est aujourd'hui éclatée entre ces deux établissements, et de faire bénéficier le gestionnaire de gares des garanties d'indépendance et des obligations de transparence et de non-discrimination dans l'accès aux facilités essentielles qui pèsent sur SNCF Réseau. C'est d'ailleurs la première option à laquelle les auteurs de la proposition de loi ont pensé.

Le rattachement à SNCF Réseau conduirait en effet à faire peser sur Gares & Connexions les contraintes d'endettement de SNCF Réseau, ce qui risquerait d'obérer ses capacités de développement des gares.

Même sous forme de filiale, un tel rattachement poserait problème, puisque, comme l'a rappelé l'ARAFER dans une étude de 2016 sur les gares, cela « ne permettrait pas de garantir une totale autonomie financière, notamment en termes de choix d'investissement, dès lors que le gestionnaire des gares serait comptablement consolidé avec SNCF Réseau ». Un rattachement à SNCF Réseau ne pourrait donc s'envisager qu'une fois la question de la dette réglée et la situation financière de SNCF Réseau assainie. Je fais d'ailleurs remarquer à cet égard que le projet de loi d'habilitation à recourir à des ordonnances du Gouvernement ne comporte aucun article relatif à la dette. Pour toutes ces raisons, il est préférable d'en rester à la solution retenue dans la proposition de loi, à savoir créer une troisième entité, filiale de l'EPIC SNCF, ce qui conférera à Gares & Connexions une véritable autonomie financière et organisationnelle. La commission est donc défavorable

remis au Premier ministre le 15 février dernier. Les auteurs de la proposition de loi ont fait le choix de transformer Gares & Connexions en société anonyme et de la rattacher à l'EPIC de tête SNCF. Nous pensons, pour notre part, qu'un rattachement à SNCF Réseau serait plus pertinent, entité soit délestée d'une part importante de sa dette. Toutefois, si le dispositif proposé par les auteurs du présent texte devait être retenu, il nous semblerait essentiel de prévenir toute future privatisation de cette structure, d'autant que les biens immobiliers de Gares & Connexions relevant de son domaine public seront déclassés et lui seront attribués en pleine propriété. Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit que le capital de la nouvelle société anonyme soit exclusivement public.

La proposition de loi prévoit que l'État demeure, quoi qu'il arrive, l'actionnaire majoritaire de Gares & Connexions, ce qui empêchera toute privatisation, sauf à passer par la loi, et donc à obtenir l'autorisation du Parlement. Ouvrir à d'autres investisseurs, publics ou privés, le capital des gares permettra de diversifier les sources de financement et favorisera le développement et la modernisation des gares, sans recourir à l'endettement. Dans son étude de 2016 sur les gares, l'ARAFER souligne à juste titre que l'ouverture du capital de Gares & Connexions à des investisseurs tiers, en premier lieu les régions, « pourrait inciter à orienter la gestion vers davantage de rigueur économique, tout en procurant à cette activité de nouvelles ressources,

qui devra être signé entre l'État et Gares & Connexions, la proposition de loi prévoyant par ailleurs que le contrat soit renouvelé tous les trois ans. Retenir une durée de dix ans me paraît utile, puisque cela permet de projeter une stratégie de développement des gares dans le long terme et de fixer des objectifs en matière d'amélioration de l'accueil en gares et de qualité de service. Cette durée a en outre été retenue par cohérence avec ce qui se pratique au sein du groupe public ferroviaire, puisque c'est également la durée de la contractualisation avec l'État

transports des données nécessaires à l'organisation des services de transport ferroviaire. Il est en effet indispensable que les autorités organisatrices de transports puissent disposer de toutes les informations utiles pour préparer et gérer les contrats de service public relatifs à l'exploitation des services ferroviaires.

du Gouvernement ? Je veux confirmer que c'est non pas seulement le gestionnaire d'infrastructures, mais bien tous les gestionnaires d'installations de services qui devront fournir des informations dans la perspective de la préparation des appels d'offres.

opérant sur le réseau ferré national devraient pouvoir faire partie du conseil d'administration de Gares & Connexions. Ils sont concernés par la situation des gares, puisqu'ils s'en serviront comme

La proposition de loi prévoit qu'au moins une des personnalités qualifiées nommées par l'État au conseil d'administration de Gares & Connexions soit un représentant des consommateurs ou des usagers, comme c'est le cas actuellement pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

mes chers collègues, nous nous opposons au déclassement des biens de Gares & Connexions lié au changement de statut et au passage en société anonyme. Nous considérons en effet que ce déclassement va permettre la vente rapide de ces biens. Dans un contexte d'austérité budgétaire et de recherche d'économies à tous crins, il est fort probable que ce déclassement tombe comme une aubaine pour les actionnaires de cette société, en l'occurrence, pour l'instant, Ainsi, l'accord de l'État, qui est prévu, est purement formel, puisque celui-ci sera à la fois juge et partie. Va-t-on brader le patrimoine des 3 000 gares présentes sur le territoire national ? À l'inverse, nous pensons que le domaine public ferroviaire doit être considéré avec la plus grande précaution, puisqu'il est support du service public, et que sa cession doit être utilisée très exceptionnellement pour des projets qui répondent eux-mêmes qui répondent eux-mêmes à l'intérêt général. Telles qu'elles sont rédigées, les dispositions proposées au titre de cet article ne prévoient aucun garde-fou à ces cessions par une entreprise publique devenue société anonyme. Nous proposons donc leur suppression. Quel ? Cet amendement vise à supprimer les dispositions de la proposition de loi relatives à la gestion domaniale de biens de Gares & Connexions qui prévoient notamment le déclassement des biens immobiliers relevant de son domaine public. Or ces dispositions ne visent que les biens immobiliers qui sont la propriété du gestionnaire des gares, et non les gares elles-mêmes, qui sont la propriété de l'État ou d'autres personnes publiques. Il s'agit en réalité de donner à Gares & Connexions la possibilité de gérer certains biens immobiliers qui servent à ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple les immeubles de bureau. La proposition de loi prévoit par ailleurs que l'État puisse s'opposer à la cession de tels biens. La commission

continuer à accentuer la séparation entre les biens de SNCF Réseau et les biens de Gares & Connexions, aujourd'hui rattachés à SNCF Mobilités. Je pense en effet que l'idée d'un déclassement pose vraiment des questions

M. Pierre Ouzoulias. Madame la ministre, nous continuons à argumenter contre votre volonté de changer le statut de Gares & Connexions. Il nous semble que certaines dispositions du présent article sont contestables et dangereuses ; nous souhaitons

relatif au transfert du personnel qui assure des prestations de services en gare, pour ensuite préciser que, à défaut d'accord dans un délai d'un an, les modalités de ce transfert sont définies par voie réglementaire.

Nous estimons donc qu'elle porte atteinte à la démocratie sociale et crée des conditions très défavorables pour les salariés. Pour cette raison, nous demandons la suppression de cette disposition. L'amendement n°

? L'amendement n° 24 vise à supprimer le renvoi à un accord entre Gares & Connexions et SNCF Mobilités du soin d'organiser le transfert des personnels de SNCF Mobilités qui assurent des prestations en gare. Or un tel accord est nécessaire afin que Gares & Connexions dispose des ressources humaines suffisantes pour accomplir sa mission.

l'article 11 prévoit qu'un accord doit être conclu entre Gares & Connexions et SNCF Mobilités, relatif au transfert des personnels assurant des prestations en gare. À défaut d'un tel accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, les modalités de ce transfert seraient arrêtées par le Gouvernement.

? Cet amendement vise à imposer aux entreprises ferroviaires de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets. Dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, nous proposerons de généraliser l'ouverture des données en temps réel à l'ensemble des services de mobilité ; nous proposerons également de donner aux autorités organisatrices la possibilité d'avoir accès aux services numériques d'achat et de réservation des services de mobilités qui sont de leur ressort territorial.

on peut difficilement demander à un service de billetterie de la SNCF de vendre les billets de ses concurrents, d'autant plus que les règles commerciales devraient conduire les uns et les autres à se distinguer par les services qu'ils offrent à leurs clients.

Cet amendement vise à garantir l'accès aux données brutes du système commun d'information des voyageurs pour les distributeurs de billets, qu'ils soient liés ou non aux entreprises ferroviaires. Cet accès permettrait à l'ensemble des distributeurs d'informer leurs clients français et internationaux en temps réel et de manière efficace.

Cet amendement vise à donner aux distributeurs de billets l'accès à « toutes données brutes » du système commun d'information et de vente de billets, ce qui me semble excessif : certaines données, par exemple les données personnelles concernant les voyageurs, n'ont pas à être transmises aux distributeurs de billets. L'obligation posée me semble donc insuffisamment définie. Par ailleurs, je rappelle que les conditions précises de la mise en place de ce système commun seront définies par un décret en Conseil d'État, pris après

que le système ferroviaire français se réorganise autour de SNCF Réseau, garant de la modernisation et de la performance des services ferroviaires. Ce rattachement accordera autonomie décisionnelle, juridique, financière et opérationnelle à Gares & Connexions.

comme l'employeur des salariés de Gares & Connexions et comme responsable de la politique de ressources humaines et des négociations sociales. Dès lors, SNCF Réseau doit percevoir un dividende sur le résultat de Gares & Connexions pour effectuer ces missions.

lorsqu'il existe des sommes distribuables. Ce dividende peut ensuite être reversé à SNCF Réseau sous forme de dotations. L'article 15 de la proposition de loi entend pérenniser ce dispositif après que Gares & Connexions aura été séparée de SNCF Mobilités et transformée en société anonyme, afin d'éviter que les dividendes issus de l'activité des gares ne soient captés en totalité par l'État et afin de faire en sorte qu'ils puissent être reversés à SNCF Réseau en vue de participer à l'entretien du réseau ferré. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État a recommandé de préciser explicitement dans la loi que ces dividendes seront reversés à SNCF Réseau en vue de l'amélioration du réseau. Tel est l'objet de cet amendement.

qui font craindre qu'un rattachement de Gares & Connexions à SNCF Réseau ne conduise à un sous-investissement dans les gares en raison du montant de la dette du gestionnaire de réseau. Pour les

pour explication de vote. La proposition de loi que nous venons d'examiner inaugure la course, contre la montre et au pas de charge, engagée par la majorité sénatoriale et le Gouvernement pour l'ouverture à la concurrence et les changements de statut au sein de l'entreprise publique SNCF. Nous souhaitons faire entendre une autre voix dans ce concert libéral qui crée de grands dangers pour le service public ferroviaire, que ce soit en termes d'offre pour les usagers, de sécurité, de couverture de l'ensemble du territoire ou encore de tarification. Après la téléphonie, l'énergie, le fret ferroviaire, ce sont maintenant les transports ferroviaires de voyageurs qui sont visés par la libéralisation, afin de permettre aux entreprises privées de faire des profits. Nous nous opposons à cette logique et portons un tout autre projet-

ans après la création de la SNCF, la question reste la même : quelle place donne-t-on au rail ? À nos yeux, le chemin de fer reste un outil puissant de désenclavement des territoires ; il est le lien entre les territoires et les hommes, un élément de la promesse d'égalité chère à nos concitoyens. Par ailleurs, voulons-nous toujours plus de camions sur nos routes et toujours plus de bus sur les axes auparavant desservis par des lignes de trains ? Ce modèle libéral, qui est celui du laisser-faire, du désengagement public, donc de la casse de l'outil industriel, préparant la concurrence, n'est écologiquement pas soutenable pour les générations futures. Le train relève de l'intérêt général et nécessite un système d'exploitation unifié, sur un réseau unique, pour garantir une offre cohérente et performante et une péréquation à l'échelle nationale.

le serons aussi au changement de statut de l'entreprise historique, prélude, comme à chaque fois, à la privatisation et à la soumission aux impératifs des marchés financiers, contre l'intérêt des citoyens. Opposants, enfin, nous le serons à la suppression du statut des cheminots, qui ouvre le piège du « tous contre tous ». ». Opposants, donc, mais également, comme nous l'avons montré hier et aujourd'hui, acteurs du débat : nous saurons être force de proposition. La

sait le ras-le-bol des usagers du quotidien concernant le TER. Et nous attendons, dans la région Hauts-de-France, une concurrence dès que possible. Pas en 2023, madame la ministre : dès 2020 si possible

les externalités positives. Je crains d'en apprendre plus demain dans la presse, puisque vous allez révéler, je crois, une étape des concertations menées

et d'offrir tous les atouts à la SNCF dans le nouveau contexte de la concurrence, ce qui nécessite en particulier de lui donner une trajectoire financière durablement équilibrée. Il est aussi nécessaire de rassurer les cheminots sur leur avenir. sur leur avenir. Je salue la qualité du travail de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, de son président, Hervé Maurey, et votre ancien collègue Louis Nègre. Je me réjouis également de la qualité des débats que nous avons eus pendant ces deux jours.

des concertations et discussions que je mène actuellement. Je le redis, l'intention du Gouvernement n'est pas d'éluder le débat devant le Parlement. Dès lors que les concertations auront suffisamment avancé, les

démarche d'ensemble pour refonder notre politique de mobilités, notamment dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités et de son volet loi de programmation des infrastructures, sur lequel nous avons débattu hier après-midi, à partir des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. La parole

Le scrutin est ouvert.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

Débat sur « la constitutionnalisation de l'IVG ». Débat sur « la politique de fret ferroviaire en France à la suite de la présentation du Rapport du Conseil d'orientation des infrastructures du 1 février 2018 ». Personne ne